La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 14 juin 2018 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, à l'été 2024, la France aura l'honneur d'accueillir les jeux Olympiques d'été, mais également, à leur suite, les jeux Paralympiques. Cet événement sportif majeur constituera un moment de joie collective. Chacun doit pouvoir y participer. Nous devons être donc en capacité de permettre à toutes et à tous de se déplacer dans de bonnes conditions. Madame la secrétaire d'État, vous le savez, seulement 3 % des stations du réseau métropolitain parisien sont aujourd'hui accessibles aux personnes à mobilité réduite. Or, pour le moment, rien n'est prévu pour modifier réellement cette situation. Bien sûr, je n'ignore pas les efforts réalisés par la RATP, en particulier pour la signalisation à destination des déficients visuels et l'accompagnement des personnes en situation de handicap mental, tout comme je me réjouis qu'aujourd'hui, enfin, la quasi-totalité des stations de RER soient accessibles et que le réseau de surface- bus, tramway -soit aménagé. De la même manière, la garantie que chaque nouvelle station, en prolongement des lignes existantes ou dans le cadre du Grand Paris Express, soit accessible est à saluer, mais on ne peut en rester là. Il faut aller plus loin et agir sur le réseau métropolitain historique. J'entends, bien entendu, les contraintes techniques, et même financières, estimées à plusieurs milliards d'euros, que pourraient engendrer des travaux d'une telle envergure. Nous ne pouvons pas réclamer l'impossible, mais nous ne pouvons pas non plus justifier d'exclure une partie de la population de notre réseau de transports en commun souterrain, dont nous faisons, à juste titre, une fierté nationale pour son efficacité et sa rapidité. Inspirons-nous de l'exemple de Londres, qui va investir plus de 200 millions de livres pour l'accessibilité de son métro ; profitons de l'accueil des jeux Olympiques et Paralympiques pour accélérer le mouvement, développer une cohérence de transports et travailler sur les noeuds intermodaux. Il serait inacceptable que nous ne nous donnions pas collectivement les moyens de faire de l'égalité une réalité dans notre capitale, à l'heure où le monde entier aura les yeux braqués sur nous. Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous nous indiquer quelle est votre ambition en la matière ? Quelles mesures comptez-vous prendre pour atteindre cet objectif collectif et combler enfin le tragique retard dont souffre notre pays en matière d'accessibilité des personnes en situation de handicap au réseau de transports en commun ? La parole est à Mme la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénatrices et sénateurs, monsieur le sénateur Jomier, le réseau de transports en commun francilien est, fort heureusement, d'ores et déjà largement accessible aux personnes à mobilité réduite. Vous l'avez rappelé, la majorité des bus parisiens le sont, tout comme 200 lignes franciliennes, soit plus de 70 % du réseau des bus de banlieue, l'ensemble des lignes de tramway et 63 gares RER. Enfin, la moitié des 375 gares SNCF franciliennes, représentant 95 % du trafic total, sont ou seront accessibles en 2024. Pour autant, vous avez totalement raison, en dehors des stations de métro récentes, toutes accessibles, celles du métro historique ne le sont pas. Elles présentent en effet une série de difficultés qui ont conduit le législateur de 2005 à les exempter largement de l'obligation de mise en accessibilité, à condition que des transports de substitution soient mis en place. C'est sur cette base qu'Île-de-France Mobilités, au conseil d'administration duquel siègent plusieurs de vos collègues conseillers parisiens, a concentré ses efforts sur le réseau de bus parisien, qui a été rendu accessible en totalité et fait office de réseau de substitution. À la veille d'accueillir dans notre capitale une manifestation mondiale d'un aussi haut relief que les jeux Olympiques et Paralympiques, il reste possible de faire preuve collectivement de plus d'agilité pour progresser sur l'accessibilité d'un réseau centenaire, comme Londres a su le faire en 2012. Je reviens justement de la capitale britannique, avec Élisabeth Borne, après après plusieurs autres déplacements, pour étudier les solutions trouvées. C'est pourquoi l'article 23 de la loi du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 prévoit que les autorités organisatrices des transports concernées, dont Île-de-France Mobilités,

Avec Élisabeth Borne, nous avons saisi conjointement la présidente d'Île-de-France Mobilités pour lui faire part de la totale disponibilité des services de l'État pour avancer sur ce rapport. Je compte sur ce document pour identifier les pistes d'amélioration de l'accessibilité des transports à tous les types de handicaps, qui pourraient notamment amener à compléter ou accélérer les aménagements prévus dans les schémas directeurs d'accessibilité dans des délais compatibles avec la tenue des Jeux en 2024. Je suis, pour ma part, favorable à ce que toute proposition d'évolution du cadre réglementaire soit explorée pour faciliter la mise en accessibilité du métro parisien. Ainsi, la possibilité juridique et pratique d'une mise en accessibilité de stations stratégiques, et non de l'ensemble d'une ligne, devra être examinée, tout comme devront être aussi examinées de nouvelles modalités d'évacuation, qui devront être conformes aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Le gouvernement précédent avait décidé de lancer une procédure de révision de la tarification de l'ensemble de ces établissements et services. L'actuel gouvernement poursuit cette démarche et la feuille de route du projet SERAFIN-Personnes Handicapées a été validée pour 2018. Il a notamment acté le lancement d'une étude nationale des coûts destinée à « appréhender les relations entre les besoins, les accompagnements, les modes d'accueil, les caractéristiques des personnes et le coût des prises en charge ». Cette réforme, vous le savez, madame la secrétaire d'État, inquiète au plus haut point les familles, les associations, mais aussi les élus. Nombre d'entre eux, en Essonne, m'ont fait part de leur profonde préoccupation quant à la perspective de fermeture de leur institut médico-éducatif, de leur foyer d'accueil médicalisé ou encore de leur maison d'accueil spécialisée. Ils sont inquiets, parce qu'ils mesurent combien ces établissements sont indispensables pour leurs administrés. Ils sont inquiets, parce qu'ils savent que ces unités de vie offrent aux enfants handicapés non seulement un accueil et un accompagnement remarquables, mais aussi une socialisation nécessaire à leur épanouissement. L'élaboration du référentiel tarifaire pour l'allocation des ressources aux établissements et services constitue le principal motif d'insatisfaction des familles et des équipes pluridisciplinaires accompagnant les enfants handicapés. La perspective d'une réforme fondée sur la seule baisse des charges structurelles au détriment des besoins réels des personnes handicapées et des projets éducatifs personnalisés est rejetée avec force. Dans le contexte anxiogène qui caractérise toute réforme, et celle-ci en particulier, pouvez-vous m'assurer, madame la secrétaire d'État, que la prise en charge globale des personnes handicapées dans des établissements adaptés à leur handicap et à leur projet de vie ne sera pas remise en cause ? Pouvez-vous m'assurer que la réforme favorisera des parcours de vie sans rupture pour les personnes handicapées ni diminution de la qualité de l'accompagnement dont elles bénéficient aujourd'hui ? Enfin, pouvez-vous m'assurer que l'allocation des ressources aux établissements et services sociaux et médico-sociaux sera équitable et permettra à ces derniers de disposer des moyens nécessaires pour répondre à leur mission première ? La parole est à Mme la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées.

Je souhaite en premier lieu le rappeler, la transformation de ce financement est indispensable. Le constat sans concession dressé dans leur rapport par Mme Jeannet et M. Vachey en octobre 2012 reste largement Le niveau des dotations des établissements et services, qui représentent au total un peu plus de 16,5 milliards d'euros, est le fruit de l'histoire, et se traduit par de fortes iniquités entre établissements similaires. Il est donc impératif de revoir ces budgets, car il n'existe aucun lien objectif entre les modalités de l'accompagnement proposé par l'établissement ou le service, le public accueilli et le niveau du budget alloué. Je souhaite aussi vous éclairer sur le sens de ces travaux, que j'ai confirmés et que j'ai confiés à l'équipe « projet » lors de ma prise de fonction. Tout le travail de refonte de la tarification doit soutenir l'objectif politique prioritaire d'une réponse adaptée aux attentes des personnes en situation de handicap. Le financement des établissements et services doit être fondé sur l'objectivation et la liaison entre les besoins des personnes qui sont accueillies et les réponses qui leur sont apportées. Cette orientation est plus que jamais nécessaire dans le cadre de la démarche « Une réponse accompagnée pour tous », généralisée depuis le 1 janvier 2018. Au travers de cette démarche est engagée une évolution systémique de l'organisation de la réponse aux personnes handicapées afin de mieux soutenir le parcours de vie en milieu ordinaire, pour les personnes qui le souhaitent, et garantir des réponses adaptées pour tous au sein des établissements pour les autres. Le dispositif de financement rénové doit précisément apporter la souplesse nécessaire pour adapter le financement des établissements et services à la complexité de certaines situations individuelles. Je souhaite enfin vous rassurer et, à travers vous, les établissements et services, ainsi que les personnes handicapées, sur notre méthode de travail. Le projet SERAFIN-PH, comme l'ensemble des grands chantiers de réforme tarifaire du champ sanitaire, social ou médico-social, est un chantier de long terme. J'ai présidé, le 27 avril dernier, son comité de pilotage, qui a permis d'arrêter la feuille de route de l'année et le calendrier de réalisation des différents d'étude sur les modèles tarifaires ou les évolutions de financement envisageables. Nous prendrons le temps de ces travaux pour disposer de données robustes et consensuelles, comme le sont les nomenclatures arrêtées dans le cadre de la première étape de ces travaux. À ce stade, aucun choix n'a été prédéfini ni arrêté. La méthode de travail concertée et coconstruite du projet SERAFIN-PH ne vise en aucune manière à menacer la qualité des accompagnements des personnes, enfants ou adultes ; au contraire, il doit la faire progresser. Vous pouvez compter sur ma détermination, car c'est l'ADN de ma mission que de partir des personnes et de leurs besoins pour coconstruire une politique.

est à Mme Josiane Costes, auteur de la question n° 272, adressée à Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Madame la secrétaire d'État, la présence de campus universitaires délocalisés dans les villes moyennes est vitale pour le dynamisme de nos territoires, particulièrement pour ceux qui sont éloignés des grandes métropoles régionales. Les formations universitaires proposées sont indispensables pour maintenir et attirer la jeunesse et la matière grise dans des villes ou des départements fragilisés par le vieillissement de la population et la déprise démographique. De plus, les cursus mis en place répondent généralement à des demandes de formation exprimées par les entreprises locales qui éprouvent des difficultés de recrutement, ce qui permet d'assurer des emplois aux jeunes diplômés. Dans le Cantal, par exemple, les 1 300 étudiants post-bac présents à Aurillac sont une bouffée d'oxygène pour l'agglomération et le département, qui soutiennent financièrement, et de façon substantielle, la délocalisation universitaire. Les collectivités concernées souhaitent développer l'offre des formations proposées afin de mieux s'adapter encore aux demandes du tissu économique local, qui ne cessent d'évoluer, avec l'objectif d'ancrer plus fortement la présence universitaire dans leur territoire. Consciente des budgets contraints des universités, je souhaiterais, madame la secrétaire d'État, connaître la position du Gouvernement dans ce domaine, et savoir si des mesures sont envisagées pour maintenir et développer ces antennes universitaires hors des métropoles régionales, car elles sont vitales pour nos territoires. La parole

Le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation travaille à développer la visibilité des externalités positives générées par la présence d'établissements d'enseignement supérieur dans leur environnement territorial sur les plans tant social qu'économique. L'université Clermont-Auvergne est ainsi présente sur six sites différents dans la région Auvergne, ce qui permet à cette université de rayonner et de participer à l'animation économique, sociale et culturelle de l'ensemble du territoire régional. Vous citez Aurillac, mais c'est également le cas de Vichy, dans laquelle le ministère soutient l'ouverture, à la rentrée prochaine, d'un département Information-communication, option journalisme, qui sera doté de 9 postes. qui sera doté de 9 postes. Le ministère soutient également le développement de l'offre d'enseignement supérieur au-delà du périmètre universitaire en Auvergne, avec l'ouverture d'une classe préparatoire B/L au sein du lycée Ambroise-Brugière de Clermont-Ferrand pour la rentrée 2018. J'espère vous avoir rassurée sur

Madame la secrétaire d'État, je suis élue dans la Nièvre, département particulièrement et dramatiquement concerné par la baisse de démographie médicale et où les patients rencontrent désormais les plus grandes difficultés pour se faire soigner. Pour mémoire, la densité de médecins généralistes y est de 82 pour 100 000 habitants, alors qu'elle est de 96 en Bourgogne-Franche-Comté et de 104 en France. La perte de chance des patients en situation d'urgence vitale y est la plus élevée de la région Bourgogne-Franche-Comté, alors que, parallèlement, l'avenir de certains services est menacé faute, semble-t-il, de personnel soignant. l'absence d'urgentiste est la raison invoquée pour la fermeture éventuelle des urgences de nuit à l'hôpital de Clamecy, et l'absence de pédiatre pour la fermeture de la maternité de Cosne-sur-Loire. Face à cette situation, il est bien évident que les habitants et les élus de la Nièvre ne pourront pas se contenter de prendre leur mal en patience et de serrer les dents, les doigts croisés, en attendant l'arrivée promise en 2025 de médecins, espérons-le, en nombre suffisant,

plusieurs mesures immédiates pourraient être mises en oeuvre. Tout d'abord, il paraît indispensable d'ouvrir des stages de médecine générale dans la Nièvre à des étudiants des facultés de médecine de Clermont-Ferrand, de Tours et surtout de Paris, qui ne sont qu'à 200 kilomètres chacune et qui sont très fréquentées par les étudiants nivernais pour d'évidentes raisons d'accès, en transport ferroviaire notamment. Il faut ensuite permettre à des étudiants de la faculté de médecine de Dijon de suivre une partie de leur cursus à l'hôpital de Nevers, selon l'ancien modèle des hôpitaux périphériques,

au sens où le prévoit l'arrêté du 18 octobre 2017, ce qui faciliterait grandement la réalisation de stages en médecine ambulatoire en milieu rural profond. Je vous demande, en conséquence, madame la secrétaire d'État, de bien vouloir m'indiquer si le Gouvernement entend faire explorer ces pistes d'évolution concrètes

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Nadia Sollogoub, votre question pose le sujet du lien entre la carte des formations en santé et la lutte contre les déserts médicaux. Vous l'avez rappelé, il n'existe pas de dispositif indiscutable permettant de fixer les professionnels de la santé dans la région dans laquelle ils ont été formés. Cette problématique appelle bien évidemment une démarche globale, qui doit être menée conjointement par l'État et les collectivités territoriales concernées. À cette fin, et s'agissant du volet « formation », plusieurs dispositifs sont mis en oeuvre.

élément essentiel d'égalité des chances de réussite. La réflexion en cours dans le cadre de la stratégie de transformation du système de santé inclut une réflexion sur l'admission dans les études de santé, et nous aurons la préoccupation qu'une offre de proximité soit proposée à tous les lycéens pour leur permettre d'accéder à ces études quel que soit leur territoire d'origine. S'agissant des stages de médecine générale, il apparaît qu'ils sont actuellement rattachés à une faculté de médecine, en fonction du découpage territorial. Cela permet l'inclusion des maîtres de stage de médecine générale dans la dynamique pédagogique de l'université, ainsi que la gestion de la répartition des étudiants par les ARS, les agences régionales de santé. Néanmoins, les élus de plusieurs territoires, situés plus loin de leur ville universitaire de rattachement que d'une autre ville ayant une faculté de médecine, ont fait part des difficultés que cela engendre pour développer des stages de médecine générale. Un travail est donc en cours avec le ministère des solidarités et de la santé pour voir comment la règle pourrait être assouplie sans pour autant complexifier l'ensemble du dispositif. S'agissant du modèle des hôpitaux périphériques, cette disposition existe toujours pour les stages d'interne. L'évolution de la formation de second cycle permet d'accroître les temps de stage hors des CHU, qu'ils soient effectués en hôpital périphérique ou en médecine générale. L'accent est également mis sur la nécessité que le service sanitaire qui se met en place atteigne prioritairement les territoires en difficulté d'accès à la prévention. En lien avec les collectivités territoriales, nous souhaitons orienter l'ensemble de la formation des professionnels de santé, notamment des médecins, vers une plus grande part d'activité hors CHU, et construire les conditions permettant de découvrir et d'adopter des modes d'exercice répondant aux besoins de la population. Des initiatives comme le dispositif Ambition PACES en région Centre, comme les antennes délocalisées de Pau ou du Havre, comme les internats ruraux développés en Aveyron, comme le recrutement de maîtres de stage en Mayenne, montrent que c'est possible. Nous avons l'ambition que les réformes à venir, tant de l'entrée dans les études de santé que du second cycle, facilitent ces dispositifs. Les services du ministère de l'enseignement supérieur, ainsi que ceux du ministère des solidarités et de la santé, sont à la disposition des élus, à votre disposition, donc, pour examiner les projets existants ou en gestation dans votre territoire. La parole

Ford, Pages jaunes, Carrefour. À côté de cela, on a des scandales financiers, des dividendes versés aux actionnaires à des taux record

Bruno Le Maire, retenu, m'a demandé de bien vouloir répondre à sa place à la question que vous posez sur l'externalisation des activités de « service clients » par le groupe Engie, dont l'État est actionnaire de référence, comme vous l'avez rappelé. Avant de vous répondre sur le fond, je veux d'abord vous faire savoir que l'État est attentif à la dimension sociale de la transformation en cours du groupe Engie. Il faut signaler à cet égard que le groupe a signé, en avril 2016, avec trois fédérations syndicales européennes, et conformément au dialogue social que vous appelez de vos voeux, un accord impliquant qu'une offre d'emploi au sein du groupe soit proposée à tout salarié concerné par des réorganisations. Cet accord prévoit aussi un important effort de formation pour adapter les compétences des salariés aux nouveaux besoins de l'entreprise. Sur le fond, la décision d'Engie d'externaliser une partie de son « service clients » résulte d'une intensification de la concurrence sur ces marchés, en lien avec la dérégulation des marchés de l'énergie. La perception du CICE en 2014 et en 2015, dont Engie a bénéficié- vous l'avez rappelé dans votre question -, ne doit pas faire oublier la situation difficile qu'a traversée le groupe jusqu'en 2016, à l'image de l'ensemble des énergéticiens de l'Union européenne. Pour y faire face, le groupe a engagé un plan de transformation ambitieux qui intègre un effort significatif de productivité. Concernant le cas spécifique des centres d'appels, ils sont confrontés à une exigence de plus en plus élevée de la part de la clientèle. Pour satisfaire à cette exigence, ils intègrent l'apport de nouveaux outils technologiques tels que l'intelligence artificielle. Par ailleurs, les réseaux et services de communication ont atteint un niveau de performance tel qu'il augmente considérablement la pression concurrentielle sur la filière même des centres d'appels chez Engie, et, malheureusement, ailleurs aussi. Dans ce contexte, les professionnels concernés et le Gouvernement travaillent au renforcement des atouts de nos entreprises et, plus généralement, à l'attractivité de notre pays. S'agissant en particulier des centres d'appels, cela se traduit notamment par le déploiement de réseaux et de services de télécommunications à très haut débit sur tout le territoire. Le Gouvernement attache, en outre, un intérêt particulier à ce que le dialogue entre les centres d'appels et les donneurs d'ordres comme Engie se développe pour renforcer les atouts de notre système économique national et permettre à ces centres de répondre efficacement aux besoins des entreprises et des usagers. Je reviens sur les cas

333 % pour les actionnaires, contre 1 % seulement pour les salariés ! Voilà la réalité ! Donc, je ne peux pas admettre votre réponse, monsieur le secrétaire d'État ! C'est un dumping social organisé par une entreprise dont l'État est actionnaire ! Alors que 1 200 emplois sont déjà sur le carreau,

présente aucun intérêt, sinon la rentabilité et le profit, qui ont été chiffrés à 5 millions d'euros ! Parce qu'une entreprise privée ne laisse rien, même pas les miettes, ils vont aller jusqu'au bout pour liquider l'affaire et l'emploi, et vous en serez donc complices

Je vous avais déjà interrogé, monsieur le secrétaire d'État, le 6 mars dernier, sur le sujet et vous m'aviez répondu qu'il n'était « pas possible au Gouvernement de répondre favorablement à ma demande d'exonération », car cette mesure serait prévue par une directive européenne. Vous n'aviez donc pas répondu au problème sur le fond. Et je vous avais rappelé, dans ma réplique, qu'il « suffi[rai]t d'une volonté gouvernementale » pour faire évoluer le droit européen en la matière.

la collecte des déchets, les forces armées, l'administration publique, les personnes handicapées et les ambulanciers. En effet, l'article 5 de la « directive 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité » prévoit ces dispositions. Si cela est possible pour les forces armées et l'administration publique, pourquoi une demande pour les sapeurs-pompiers dans le cadre de leurs interventions serait-elle refusée par l'Union européenne ? Cette demande est justifiée. Monsieur le secrétaire d'État, l'article 19 de la directive permet d'autoriser un État membre à introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires pour des raisons de politique spécifiques. votre réponse du 6 mars dernier n'est donc pas satisfaisante. Aussi, je vous demande, monsieur le secrétaire d'État, si le Gouvernement entend avoir enfin la volonté politique de demander à Bruxelles d'introduire une exonération de la TICPE sur le carburant consommé par les sapeurs-pompiers dans le cadre de leurs missions.

tout d'abord, souligner que le Gouvernement partage l'objectif d'alléger autant que possible les charges qui pèsent de manière générale sur les services départementaux d'incendie et de secours, compte tenu de leur apport fondamental à l'intérêt général et à la solidarité nationale. C'est dans ce sens que travaille le ministre d'État, ministre de l'intérieur, en prenant notamment des mesures spécifiques

qui restreint les marges de manoeuvre des États. Peut-être votre question va-t-elle me permettre de préciser la réponse que je vous avais faite le 6 mars dernier. Au titre de cette directive, d'une part, l'article 5 permet uniquement d'appliquer un tarif réduit de taxes aux administrations publiques ou aux forces armées, sans pouvoir aller jusqu'à une exonération. D'autre part, l'article 19 de ce même texte, que vous avez cité, permet aux États membres d'introduire auprès de la Commission une demande particulière pour abaisser les tarifs de l'accise ou obtenir une exonération à certaines conditions : d'abord, que cette demande s'inscrive dans le cadre d'une politique spécifique que la Commission fasse une proposition au Conseil- ce que vous n'avez pas rappelé ; enfin, que le Conseil l'adopte à l'unanimité, et nous savons, les uns et les autres, l'immense difficulté qu'il y a à obtenir l'unanimité sur des considérations fiscales. En outre, il s'agit d'une procédure très longue, qui ne permettrait d'obtenir qu'une dérogation temporaire. C'est pour ces raisons que la France a fait le choix de ne pas transposer, depuis 2003, la faculté prévue à l'article 5 ni d'actionner la procédure prévue à l'article 19. Il s'ensuit qu'aucune structure publique, quelle que soit l'importance de sa contribution à la solidarité nationale, ne peut bénéficier, aujourd'hui, d'un régime particulier au regard de la TICPE. Sans méconnaître l'importance et la difficulté des missions dont les SDIS ont la charge, le recours à un tarif réduit de TICPE pour les consommations de ces seuls services ne serait pas justifié au regard du régime de TICPE des consommations de l'ensemble des autres administrations publiques supportant ces impôts, y compris les forces de police et les forces armées. Votre proposition serait en effet dérogatoire par rapport à ce dispositif déjà réduit dont les uns et les autres disposent. J'ajoute encore que la recette de TICPE est en partie affectée aux départements et qu'il ne paraît pas opportun, de manière au moins conjoncturelle, alors qu'une réflexion globale est en cours sur le financement des collectivités territoriales, d'introduire une exonération ciblée supplémentaire qui ne manquerait pas d'appeler de nombreuses demandes similaires, au risque de perturber le modèle de financement des collectivités. En outre, nous souhaitons que le financement des SDIS puisse être abordé sous l'angle de l'appréciation des ressources qui leur sont allouées- cela renvoie à mes premiers mots. Je pense notamment au plan que le ministre d'État, ministre de l'intérieur met en place pour mieux financer et soutenir SDIS. Cela renvoie aussi aux discussions que le Gouvernement mène actuellement avec l'Assemblée des départements de France pour faire en sorte de permettre aux départements de mieux faire face aux besoins dans ce domaine, comme dans d'autres.

le répète : si le Gouvernement veut faire avancer ce dossier, il peut le faire, même si c'est long ! On commence aujourd'hui et on se donne les moyens de suivre ce dossier au plus haut niveau à Bruxelles, et je suis sûre qu'on peut y arriver tous ensemble

l'insuffisance des effectifs de ce même commissariat. En retour et pour seule réponse, le ministre d'État, ministre de l'intérieur m'indiquait qu'il demandait à la direction générale de la police nationale de faire un point précis sur la situation signalée. Et depuis un an, plus rien, plus de nouvelles sur ce dossier. Quelle est donc la situation de ce commissariat ? En 2015, il comptait 96 membres du corps d'encadrement et d'application actifs, CEA, et 16 adjoints de sécurité. En 2018, on ne compte plus que 91 membres du CEA et 11 adjoints de sécurité. Bilan : 10 effectifs en moins ! Or dans le même temps, ou presque, le territoire de compétence du commissariat a été élargi considérablement à d'autres quartiers, comme Baliste, Malvézy, Amarats, Crabit et aux zones La Nautique et Cap de Pla Toujours dans le même temps, la même zone de police voyait sa démographie augmenter de près de 2 500 habitants. Et toujours dans le même temps, la délinquance de plus en plus violente était en hausse, comme l'atteste le classement

Plus grave, ces locaux ne sont même pas sécurisés, ce qui explique qu'un Narbonnais, en avril dernier, alors que sa garde à vue prenait fin, se soit défenestré depuis le troisième étage.

Qu'en pense le Secrétariat général pour l'administration du ministère à Marseille qui a, semble-t-il, le dossier complet en main ? Que compte dire M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur à la direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières ? Ces fonds ont été annoncés, madame la secrétaire d'État. L'État doit donc

qui ne pouvait être là ce matin. Les policiers travaillent au quotidien avec courage et un sens élevé de l'intérêt général, vous l'avez dit. Dans un contexte de plus en plus difficile et violent, ils sont là pour faire appliquer les lois et protéger les Français. Leurs conditions de travail sont, bien sûr, un sujet essentiel pour le ministre de l'intérieur, comme plus largement la nécessité de leur garantir les moyens d'accomplir leurs missions dans les meilleures conditions d'efficacité et de sécurité. Cette priorité se traduit concrètement. présentée le 24 janvier dernier une programmation immobilière ambitieuse pour la police nationale et pour la gendarmerie nationale, qui s'appuie sur des budgets accrus. La police nationale est ainsi dotée d'un budget « immobilier » de 196 millions d'euros par an au titre de la programmation triennale, soit 5 % de plus par rapport à 2017. Autre paramètre important, en 2018, 45 millions d'euros de crédits- au titre des crédits TATE, travaux d'aménagement et d'entretien -sont déconcentrés aux responsables locaux pour des travaux d'aménagement et d'entretien courant, contre 19 millions d'euros en 2016. Il traduit un choix de confiance et d'efficacité. Ces initiatives portées localement permettront de mettre en oeuvre ces moyens. Les besoins immobiliers sont cependant très nombreux et malgré des efforts budgétaires, tout ne peut être accompli de façon immédiate. S'agissant du commissariat de Narbonne, des avancées ont été enregistrées.

acquisitions diverses et film de protection visuelle, en particulier. Bien sûr, il y a encore à faire. D'importants projets sont programmés, notamment la restructuration des locaux du rez-de-chaussée et l'optimisation de surfaces afin de pallier des problèmes d'insalubrité, de confidentialité et de sécurité.

Cet effectif devrait rester stable dans les mois à venir. L'effectif prévu au 31 octobre 2018 s'établit en effet à 128. Je tiens à ajouter que cette circonscription de police bénéficie d'un nombre de gradés et de gardiens de la paix, qui représente, vous le savez, l'essentiel des policiers présents sur la voie publique,

sur ma faim ! Vous avancez des crédits pour des études en cours, mais vous ne répondez pas à ma question : que sont devenus les 900 000 euros qui nous ont été annoncés en 2016 ?

je vous demanderai, madame la secrétaire d'État, de transmettre à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur la proposition avancée par un syndicat visant la mise en place d'un système dit « de vacation forte », avec l'octroi d'un week-end sur deux pour les fonctionnaires intervenant sur la voie publique en police secours, au lieu de 1 pour 6 actuellement. Il paraît que ce système permet de cumuler plusieurs groupes qui se chevauchent sur un temps donné, chose qui a été refusée par le ministère de l'intérieur pour Narbonne, alors qu'il fonctionne notamment à Perpignan, à Toulouse et à Nîmes. La parole est à M.

que l'ONERA annonce son déménagement ! Voilà plus de vingt ans que des études sont faites année après année, chaque fois qu'un président est nommé- tous les quatre ans ! Voilà plus de vingt ans qu'on attend une décision

Au moment où, madame la secrétaire d'État, on recherche des financements- ils sont indispensables, ne serait-ce que pour l'ONERA et son déménagement -, au moment où le Gouvernement, après d'autres, annonce vouloir rechercher du foncier en région parisienne pour construire, toutes les conditions sont réunies afin qu'une décision soit prise. Ma question est simple, madame la secrétaire d'État : pouvez-vous me confirmer le déménagement de l'ONERA ? Pouvez-vous en préciser le calendrier

a été signé le 14 décembre 2016. L'ONERA est actuellement implanté sur huit sites en métropole. En ce qui concerne l'Île-de-France, le COP prévoit effectivement la cession des deux emprises de Meudon et Châtillon en vue de regrouper tous les services de l'Office sur le site de Palaiseau. Les sites actuels d'Île-de-France, situés à Meudon, Châtillon et Palaiseau, comptent environ 1 200 personnes, soit plus de 60 % des personnels de l'Office. Ce regroupement à Palaiseau doit notamment permettre à la fois un fonctionnement intégré des différents départements de l'ONERA et, bien sûr, des économies de fonctionnement.

Plus globalement, la logique de ce regroupement à Palaiseau procède aussi de la proximité du potentiel scientifique unique en France qui se trouve autour du plateau de Saclay. On peut comprendre la complémentarité entre l'ONERA et ce potentiel scientifique. L'opération de regroupement doit être financée, pour l'essentiel, par le produit de cession des emprises de Châtillon et Meudon. Un plan de financement est actuellement à l'étude, fondé, en particulier, sur un prêt de la Banque européenne d'investissement, la BEI, afin de pouvoir lancer ce projet sans faire appel à la mobilisation de crédits budgétaires. L'opération devra ensuite être validée par les instances requises, notamment en conseil d'administration. Une fois lancée, la durée totale de l'opération de regroupement est estimée à cinq ans.

On connaît tout cela. Ce qui est attendu maintenant, madame la secrétaire d'État, c'est une décision. Le jour où une décision intervient, l'ONERA s'adaptera, les administrations aussi. Pour ce qui est de Meudon,

qui mette un terme aux tergiversations des diverses administrations concernées. Le lieu d'implantation, Palaiseau, est connu depuis déjà pas mal d'années et les données du dossier sont connues de tous. Je sais,

de la Charte européenne des langues minoritaires et régionales. Certes, la décision du Conseil constitutionnel en date du 15 juin 1999 considère que ce texte était inconstitutionnel parce qu'il portait atteinte aux articles 1et 2 de la Constitution, disposant que la République est indivisible et que sa langue est le français. Ces principes interdisent qu'il soit reconnu des droits, par exemple, linguistiques, à un groupe humain identifié et distinct du corps national indivisible. Il ne peut exister des droits propres à certaines communautés. Toutefois, je fais le constat que l'enseignement bilingue existe au pays basque, en Bretagne, en Corse, en Occitanie, en Alsace, au pays catalan et en outre-mer. L'enseignement du flamand occidental a pris du retard, selon ses défenseurs. Ces derniers ont lancé des actions afin de déclencher, de la part des pouvoirs publics, un certain nombre d'initiatives. En 2007, une expérimentation de l'enseignement du flamand occidental a été lancée dans six écoles de la région Hauts-de-France, mais l'initiative ne s'est pas étendue. Or, selon le code de l'éducation, la durée maximale d'une telle initiative est de cinq ans. En réalité, le flamand occidental ne serait pas inscrit au registre des langues régionales du ministère de l'éducation nationale, considérant que cette langue serait assimilée au néerlandais. Néanmoins, je précise avec satisfaction que les élus de la région Hauts-de-France ont accepté de créer un office public du flamand occidental, à l'instar du breton et de l'alsacien. 70 000 euros seront accordés afin « d'accompagner les associations à la préfiguration de cet office ». Le but est de créer une structure adaptée au développement de cette langue régionale dans le domaine de la culture, de l'emploi et de l'enseignement. cet effort n'est qu'une étape aux yeux des intéressés, qui souhaitent institutionnaliser l'enseignement de cette langue dans les écoles publiques. S'il ne s'agit pas de revendiquer une langue co-officielle, je demande si, culturellement, madame la secrétaire d'État, vous entendez encourager l'apprentissage d'une langue locale, qui n'est en rien une menace à l'unité ou à l'indivisibilité de la République, mais une démarche culturelle régionale sans être une revendication régionaliste. La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des armées. des armées. Monsieur le sénateur, je vous prie d'excuser le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui m'a chargée de vous apporter une réponse ce matin.

C'est dans cet esprit qu'est examinée la situation du flamand occidental, qui peut trouver une place à l'école. En effet, l'article L. 312-11 du code du code de l'éducation dispose que les enseignants des premier et second degrés « sont autorisés à recourir aux langues régionales, dès lors qu'ils en tirent profit pour leur enseignement. Ils peuvent également s'appuyer sur des éléments de la culture régionale pour favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires et de culture et des programmes scolaires ». En outre, l'enseignement du néerlandais dont vous avez parlé, qui est une langue de communication avec la région flamande de Belgique et les Pays-Bas, est une priorité pour l'académie de Lille, notamment pour le département du Nord, aussi bien pour l'enseignement primaire que pour le collège et le lycée. L'apprentissage de cette langue répond notamment à de forts enjeux économiques et d'employabilité. De fait, c'est la connaissance de la langue néerlandaise qui permet aux élèves de la zone frontalière de trouver des débouchés professionnels de l'autre côté de la frontière, ce qui n'exclut pas, bien sûr, une connaissance de ses variations dialectales. dialectales. Ainsi, la proximité linguistique de la langue régionale flamande avec la langue néerlandaise peut être avantageusement mise à profit lors des séances consacrées à l'apprentissage de cette dernière ; un travail peut être mené sur les nuances dialectales et sur les réalités culturelles- coutumes, expressions, art -de l'espace linguistique du franco-flamand. Signalons aussi qu'un enseignement de la variante française du flamand occidental est présent dans trois écoles primaires publiques, dans le cadre d'une expérimentation. La poursuite de cette expérimentation dépendra des conclusions de l'évaluation qui sera conduite par les services de l'académie de Lille. Enfin, à l'école primaire, la sensibilisation au flamand occidental et à la culture qu'il porte peut aussi faire l'objet d'activités éducatives et culturelles complémentaires conduites durant le temps périscolaire- temps important en lien, par exemple, avec les associations locales bénéficiant d'un agrément pour intervenir en milieu scolaire. Au total, nous sommes attentifs à ce que cet apprentissage culturel perdure dans cette région.

de Cassel : « J'ai un tropisme belgo-luxembourgeois qui fait que je me sens naturellement chez moi en Flandre. C'est un coin pour lequel j'ai une tendresse toute particulière. Ici, dès mon arrivée, j'ai été en admiration face aux bâtiments de la place, remarquablement bien entretenus. Il y a également toutes ces traditions flamandes, notamment la sympathique danse des Reuze- des Reuze- les géants de notre Flandre -avec cet air entraînant et cette rythmique qui fait qu'on ne peut s'empêcher de danser. Je trouve qu'il y a un charme inouï à Cassel. Vraiment. J'espère que tous les Français tomberont sous le charme de cette cité flamande comme je l'ai été. » La parole est

de votre exploit ! Avec bon nombre de mes collègues, nous avons été très nombreux à vous alerter sur les conséquences de la diminution draconienne des crédits alloués par le Centre national pour le développement du sport, ou CNDS, au cours de l'exercice budgétaire 2018.

L'incompréhension et l'inquiétude sont grandes au sein des clubs des 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine, qui doivent faire face à une diminution de près de 50 % de leurs ressources. En outre, le caractère arbitraire d'une telle décision, annoncée sans concertation, accentue l'incompréhension légitime de l'ensemble des responsables et des dirigeants du mouvement sportif. La saison sportive est déjà bien amorcée et l'on peut se demander avec quels moyens les associations, été durement impactées par la réduction des contrats aidés, vont pouvoir mener à bien les politiques déjà engagées pour l'année en cours. Madame la ministre, vous déclarez vouloir mener une politique sportive ambitieuse, qui nous ferait passer d'une nation de sportifs à une nation sportive. Quoi de meilleur

risquent d'exclure de nombreux territoires, tout en imposant une injuste sélectivité des projets soutenus par les associations locales, ainsi qu'une absence de reconnaissance du bénévolat ? Comment, face à de telles diminutions de moyens, parvenir à maintenir la mobilisation du mouvement sportif et assurer le maintien de la vie associative ? La décision récente de dégager 5,6 millions d'euros en faveur des clubs sportifs en difficulté n'est pas de nature à apaiser la colère des responsables du mouvement sportif, tant à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine qu'à celle du Pourriez-vous, madame la ministre, nous préciser les mesures que vous comptez prendre de manière à rassurer les responsables du comité régional olympique et sportif de la Nouvelle-Aquitaine et leurs collègues du comité olympique de la Gironde, afin qu'ils puissent remplir les missions qui leur sont confiées

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Madrelle, dès 2018, j'ai souhaité clarifier les interventions menées par le ministère des sports et le CNDS. Notre action publique a besoin de cohérence et de lisibilité. Le CNDS a donc été recentré sur son coeur de métier

Pour garantir l'efficacité de l'intervention du CNDS, la part territoriale de son action doit être plus sélective. Éviter le saupoudrage et concentrer les moyens sur la résorption des inégalités territoriales, voilà l'objectif Je le crois juste et surtout nécessaire aujourd'hui, quand on sait qu'il y a encore des quartiers qui, comme pour la téléphonie mobile, n'ont aucune infrastructure sportive. Toutefois, monsieur le sénateur, j'ai entendu les difficultés que rencontrent certains petits clubs, difficultés dont les élus se sont fait le relais. C'est pourquoi une enveloppe exceptionnelle de 5,6 millions d'euros, dégagée grâce à la bonne gestion des crédits du CNDS et de la direction des sports, va être allouée dès ce mois de juin par le CNDS aux clubs en difficulté. Il appartiendra aux directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, en qualité de délégués territoriaux du CNDS, de cibler les clubs qui en ont le plus besoin, dans le cadre des commissions territoriales.

et de la santé. Madame la ministre, comme vous le savez, deux expérimentations sont en cours dans plusieurs de nos départements pour évaluer la possibilité d'un remboursement par l'assurance maladie des suivis psychologiques hors des

non médicamenteuses des troubles en santé mentale d'intensité légère à modérée chez l'adulte de 18 à 60 ans. Ce dispositif, prévu pour quatre ans, devrait permettre aux pouvoirs publics d'évaluer l'intérêt et la faisabilité d'une prise en charge par la sécurité sociale des actes des psychologues libéraux. Si je ne peux que partager cet objectif, permettez-moi, d'une part, de regretter fortement que les professionnels concernés, à savoir les psychologues, n'aient pas été associés à ces démarches et ne le soient toujours pas, malgré la lettre ouverte qu'ils vous ont adressée en janvier dernier, d'autre part, de ne pas partager les raisons qui vous poussent à soumettre ces professionnels de santé à un pilotage médical qui détermine, prescrit et contrôle les actes mêmes des psychologues. Mes remarques font écho à celles des psychologues eux-mêmes. En effet, ce procédé choque à juste titre la profession, qui y voit un acte de mépris, un manque de reconnaissance, voire une mise sous tutelle médicale. Les psychologues ne seraient-ils donc pas assez légitimes pour évaluer par eux-mêmes la souffrance psychique et proposer des solutions ?

conviendrez que le taux de remboursement proposé pour ces consultations, entre 22 et 32 euros, est bien trop bas au regard du prix d'une consultation et ne peut permettre à ces professionnels d'exercer correctement leur métier. C'est pourquoi je voudrais savoir, madame la ministre, comment vous comptez, d'une part, associer les psychologues à ces expérimentations de façon à sortir d'une vision médico-centrée de la prise en charge psychologique

Nous innovons aujourd'hui en expérimentant d'autres modalités de prise en charge. L'expérimentation Écout'Émoi vise à diminuer l'éventuelle souffrance psychique

de santé mentale, repérer plus précocement les troubles et évaluer la souffrance psychique pour prescrire, si besoin est, des consultations chez des psychologues cliniciens libéraux à des jeunes en situation de mal-être ne présentant pas de troubles sévères. Ces consultations seront prises en charge par l'assurance maladie dans le cadre de l'expérimentation. Pour des troubles plus importants, les psychiatres resteront en première ligne. Tous les professionnels au contact des jeunes seront impliqués dans ces expérimentations, qu'il s'agisse des professionnels de santé, des professionnels de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ou des maisons des adolescents, qui coordonneront le dispositif sur le terrain. Cette expérimentation sera menée en Île-de-France, dans le Grand Est et dans les Pays de la Loire. Une seconde expérimentation est portée par l'assurance maladie en Haute-Garonne, dans le Morbihan et dans les Bouches-du-Rhône. Elle porte sur la prise en charge des thérapies non médicamenteuses en médecine de ville pour les troubles en santé mentale d'intensité légère à modérée. Elle s'adresse aux adultes de 18 à 60 ans souffrant de trouble dépressif ou anxieux, de trouble de l'adaptation, d'intensité légère à modérée, ou de syndrome médical inexpliqué. Cette expérimentation propose aux patients de mener, après évaluation par un médecin, des séances de psychothérapie avec un psychologue clinicien ou un psychothérapeute ; ces séances seront prises en charge par l'assurance maladie dans le cadre du Ces deux dispositifs expérimentaux vont faire l'objet d'évaluations scientifiques avec l'ensemble des acteurs impliqués ; les résultats de ces évaluations permettront d'élaborer des recommandations en cas de généralisation.

tout comme leur autonomie, d'ailleurs. Aujourd'hui, l'âge moyen d'entrée en établissement est de 87,16 ans, ce qui amène inévitablement une dépendance marquée des résidents et une hausse nécessaire du temps qu'il faut consacrer à chacun d'eux. Madame la ministre, afin d'assurer la bientraitance de nos aînés, il faut des moyens importants en personnel et en équipement. Or les budgets des EHPAD sont sans cesse affectés par les baisses des dotations octroyées par l'Agence régionale de santé, l'ARS, du fait de la nouvelle réforme de la tarification, et ce alors que les budgets de fonctionnement sont déjà réduits au strict nécessaire. En conséquence, les besoins des résidents ne peuvent être correctement satisfaits et les structures ne peuvent être entretenues comme elles le devraient.

découle des conditions réglementaires nécessaires pour occuper un tel poste : le niveau de connaissances et d'aptitude requis est tel que les candidats, une fois admis et formés, sélectionnent des postes dans des établissements de taille importante et en zone urbaine, délaissant malheureusement ceux, de taille modeste, qui sont implantés dans les zones rurales. Face à cette absence de moyens, les personnels des EHPAD se sont mis en grève à deux reprises, le 30 janvier et le 15 mars derniers. En réponse, madame la ministre, vous avez annoncé, au mois d'avril, vouloir aboutir d'ici à l'automne à un ajustement de la réforme controversée du financement des EHPAD. Vous avez également confirmé une mesure financière : la neutralisation, pour les années 2018 et 2019, des effets de baisse de recettes au titre de la dépendance. Madame la ministre,

avait été engagée avant mon arrivée au ministère ; j'ai rapidement nommé un médiateur, M. Pierre Ricordeau, pour examiner précisément la situation. Des travaux vont désormais s'engager, avec les fédérations représentant les EHPAD et l'Assemblée des départements de France, pour permettre aux départements de fixer un tarif « dépendance » plus adapté aux besoins des EHPAD de leur territoire. La montée en charge de la réforme de la tarification des soins dans les EHPAD, issue de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, qui permet d'augmenter, en moyenne, les financements alloués aux soins, était prévue jusqu'en 2023. Afin de renforcer plus rapidement la présence de personnels soignants au sein des EHPAD, j'ai demandé à ce que l'ensemble des établissements atteignent leurs nouveaux tarifs cibles beaucoup plus rapidement, d'ici à la fin de l'année 2021. Cela représente un effort supplémentaire de 143 millions d'euros, qui s'ajoutent aux 217 millions d'euros qui étaient déjà prévus sur cette période pour le recrutement de personnels soignants dans ces établissements. Dans le Dans le Puy-de-Dôme, comme cela a été indiqué dans l'instruction budgétaire nationale du 15 mai 2018, un mécanisme a été instauré cette année pour neutraliser,

11 EHPAD, seront intégralement compensées cette année en crédits non reconductibles ; quant aux convergences négatives « dépendance », l'ARS va notifier, en plus des crédits non reconductibles pour tous les EHPAD du Puy-de-Dôme, 248 795 euros pour les 32 établissements concernés. Je vous remercie,

Madame la ministre, ma question porte sur le fonctionnement de la société commerciale MédecinDirect. La télémédecine s'implante dans le paysage médical français, ce qui est une très bonne chose. Toutefois, le fonctionnement de la société MédecinDirect m'a alertée. Cette société revendique 1 600 téléconsultations par mois. Des médecins y sont joignables par mail ou par téléphone 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour effectuer un diagnostic et rédiger une ordonnance. L'article R. 4127-19 du code de la santé publique dispose que la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. D'autre part, la téléconsultation médicale figure à l'article R. 6316-1 de ce même code, qui précise que la téléconsultation a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient ». Selon la loi, une téléconsultation est donc une consultation à distance qui permet au professionnel de santé médical requis de réaliser une évaluation globale du patient, en vue de définir la conduite à tenir à la suite de cette téléconsultation. Or, avec MédecinDirect, le patient et le médecin s'écrivent ou se parlent, mais ils ne se voient jamais. La question se pose donc de savoir si cette société commerciale est un établissement de santé soumis à l'autorisation de l'Agence régionale de santé, Le cas échéant, madame la ministre, je souhaiterais savoir si une ARS est en mesure d'autoriser une société commerciale relevant du code de commerce à prodiguer des actes médicaux. La parole est à Mme la ministre des solidarités et de la santé. Lassarade, la société MédecinDirect a signé un contrat de télémédecine avec l'Agence régionale de santé d'Île-de-France le 14 décembre 2015 ; ce contrat a été renouvelé le 14 décembre dernier. Ses activités de télémédecine n'ont débuté qu'en septembre 2016, après l'obtention de l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. MédecinDirect est une plateforme qui permet la mise en relation par écrit, téléphone ou vidéotransmission, suivant son choix, avec un médecin pour un conseil personnalisé ou une téléconsultation. Ses principaux clients sont des assureurs complémentaires santé et des mutuelles,

n'entre pas dans le champ d'application de la télémédecine. Le contrat signé avec l'Agence régionale de santé a seulement pour objet de déterminer les objectifs et les modalités de réalisation des téléconsultations de MédecinDirect. Ce contrat permet la déclinaison des orientations régionales fixées dans le projet régional de santé : améliorer l'accessibilité de tous à des soins de qualité sur l'ensemble du territoire, consolider la permanence de soins, renforcer la prise en charge des maladies chroniques et viser au développement des usages de la téléconsultation en garantissant la qualité et la sécurité des soins. L'article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 précise que « les actes de téléconsultations remboursés par l'assurance maladie sont effectués par vidéotransmission »., la vidéotransmission n'est pas une obligation dans une téléconsultation qui n'est pas prise en charge par l'assurance maladie. Je vous confirme, enfin, que les téléconsultations de médecins directs constituent une pratique médicale soumise aux règles de l'exercice de la médecine en France, qui imposent notamment l'inscription auprès d'un conseil ordinal. La parole

à l'excellence de la téléexpertise à laquelle les Français auraient droit, la marchandisation de la santé, avec tous les excès que cela peut impliquer

Madame la ministre, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la drépanocytose, la maladie génétique la plus répandue dans le monde. L'ONU en a fait sa quatrième priorité de santé publique.

longtemps été qualifiée de « maladie des noirs », car elle a été identifiée et caractérisée en premier lieu au sein de la population afro-américaine aux États-Unis. Il est aujourd'hui admis que la mutation s'est renforcée dans les populations occupant les régions du globe soumises à une forte prévalence du paludisme. C'est pourquoi la drépanocytose, surtout présente en Afrique subsaharienne, l'est également sur le pourtour méditerranéen et en Inde, mais également, héritage du commerce triangulaire et de l'esclavagisme, sur le continent américain.

Il n'existe à ce jour pas de traitement curatif. Des traitements à l'efficacité aléatoire existent pour prévenir les crises et certains symptômes. C'est pourquoi, madame la ministre, pour une bonne prévention, pour l'éducation à la maladie, et pour qu'en cas de crise le diagnostic soit immédiatement posé, le dépistage néonatal est indispensable. En l'an 2000, la France instaurait un dépistage de la drépanocytose à la naissance sur tout son territoire. Systématique dans les outre-mer, il est ciblé dans l'Hexagone en fonction de l'origine des parents. Malheureusement, des enfants drépanocytaires naissent encore aujourd'hui sans être dépistés. Ils sont soignés et, parfois, hospitalisés plusieurs fois avant que le diagnostic soit posé. Comment pouvons-nous tolérer de laisser ces enfants dans d'immenses souffrances alors que nous disposons des moyens techniques et financiers En juillet 2009, Mme Roselyne Bachelot, alors ministre de la santé, présentait son plan Santé outre-mer. Elle déclarait alors : « Bien qu'étant la maladie génétique la plus fréquente en France, la drépanocytose n'a pas bénéficié de la même attention que d'autres maladies génétiques. Il est temps de mettre fin à cette situation en rétablissant la qualité des soins et l'égalité de tous devant la maladie. Madame la ministre, vous êtes médecin hématologue, vous connaissez donc mieux que quiconque dans cet hémicycle cette maladie, vous savez mieux que quiconque ici la souffrance des drépanocytaires. Madame la ministre, faites de la drépanocytose une grande cause nationale Systématisez le dépistage néonatal de la drépanocytose sur tout le territoire national en l'intégrant au test de Guthrie ! Madame la ministre, je ne saurais terminer mon propos sans évoquer la situation particulière de l'hôpital de Cayenne et, surtout, de ses urgentistes. Je crois savoir que se tiendra demain une réunion très importante sur une sortie de crise. J'apprécierais que toute votre attention soit portée sur cette sortie de crise.

vous avez raison, la drépanocytose est une maladie que je connais particulièrement bien et qui est grave pour les patients. Je suis heureuse de pouvoir vous rappeler toutes les actions menées aujourd'hui pour faire reculer cette maladie.

par un dépistage le plus précoce possible, afin d'éviter au maximum les complications et séquelles ainsi que l'altération de la qualité de vie des personnes. La drépanocytose fait partie aujourd'hui des cinq maladies inscrites au programme national de dépistage néonatal. En France, le dépistage de cette maladie est généralisé chez tous les nouveau-nés depuis 1989 dans les départements et régions d'outre-mer. En métropole, il n'est réalisé que depuis 1995 et seulement chez les nouveau-nés présentant un risque particulier de développer la maladie en fonction de l'origine des parents. La question de l'efficacité du dépistage néonatal ciblé de la drépanocytose en métropole n'est pas nouvelle. En 2014, la direction générale de la santé avait souhaité que la Haute Autorité de santé examine la question de l'élargissement éventuel du dépistage à l'ensemble de la population, quelle que soit l'origine des parents. Dans son rapport, cette dernière n'avait pas relevé de signaux clairs d'un manque d'efficacité de la stratégie du dépistage néonatal ciblé.

préconisé de mettre en place, à titre expérimental, un dépistage généralisé dans une région de métropole où la prévalence de la drépanocytose est élevée, par exemple l'Île-de-France, avant d'envisager une généralisation dans toute la France métropolitaine. Cette préconisation a retenu toute mon attention. C'est pourquoi j'ai décidé, notamment au regard des données médicales récentes qui m'ont été apportées, de saisir de nouveau la Haute Autorité de santé, afin qu'elle puisse indiquer si les données disponibles peuvent conduire à à une révision de son avis de 2014. Il s'agira également de définir, si tel était le cas, les modalités pertinentes d'une généralisation de ce dépistage néonatal sur tout le territoire métropolitain.

et de la santé. Madame la ministre, on constate des difficultés croissantes dans l'approvisionnement des pharmacies, y compris celles des centres hospitaliers, quand il ne s'agit pas tout simplement de ruptures de stock, pendant parfois plusieurs mois. Cette pénurie frappe aussi les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, avec une hausse des difficultés d'année en année

Parmi les causes de ces difficultés, on compte bien sûr l'explosion de la demande mondiale dans un contexte où les grands laboratoires fusionnent jusqu'à se trouver en situation de quasi-monopole dès lors, les possibilités de recours et les capacités de production baissent. De même, la dépendance au marché mondial a des effets sur la fourniture en matières premières pour les médicaments qui ne sont pratiquement plus fabriqués en France. Dans cette situation de pénurie, le laboratoire Mylan par exemple, qui produit l'antibiotique Augmentin®, d'utilisation courante à l'hôpital, a annoncé qu'il cesserait sa production à destination de la France pour se tourner vers l'export d'ici à la fin de cette année, mais qu'il resterait possible de lui acheter des antibiotiques au prix de l'export, c'est-à-dire pour un autre cas existe, celui des médicaments dérivés du sang, dont les immunoglobulines polyvalentes. L'insuffisance du stock des laboratoires LFB et CSL Behring a obligé parfois à retarder l'instauration de cures, l'ANSM demandant aux prescripteurs de hiérarchiser les indications, afin d'utiliser les stocks restants pour les indications les plus prioritaires. Cette situation conduit aussi les instances à autoriser des spécialités équivalentes destinées initialement aux marchés turc et brésilien, avec des notices qui ne sont pas en français et sans étiquette de traçabilité.

que les laboratoires respectent leurs engagements, mais également pour limiter les surcoûts pour nos hôpitaux. Nous vous demandons donc, madame la ministre, s'il n'est pas envisageable

Watrin, l'approvisionnement en médicaments est un objectif de santé publique majeur, en particulier pour les médicaments d'intérêt thérapeutique. Dans certains cas, l'indisponibilité est susceptible d'entraîner un problème de santé publique,

L'Agence générale des équipements et produits de santé, l'AGEPS, que vous mentionniez, met aujourd'hui en oeuvre la politique de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en matière d'équipements et de produits de santé. se compose de plusieurs pôles, dont le pôle Établissement pharmaceutique de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Ce dernier joue un rôle essentiel dans la recherche, le développement, la production et la mise à disposition des patients des médicaments indispensables, qui répondent à des situations rares ou à des indications orphelines. Il s'agit de situations non prises en charge par l'industrie pharmaceutique ou de médicaments nécessitant une adaptation galénique pour répondre aux besoins de populations particulières, comme les enfants et les personnes âgées. Toutefois, cet établissement pharmaceutique public n'a pas pour mission de produire des médicaments en grande quantité destinés à couvrir le marché français. Conformément à l'article R. 5124-69 du code de la santé publique, l'AGEPS ne peut fabriquer des médicaments qui disposent déjà d'une autorisation de mise sur le marché exploitée dans le secteur concurrentiel. Dès lors, l'Agence n'a pas pour mission de suppléer les laboratoires du secteur privé en cas de rupture d'approvisionnement en médicaments produits par ces derniers. Par ailleurs, la production de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur par un établissement public ne garantirait pas des ruptures liées en particulier à un problème d'approvisionnement en matières premières qui se situe le plus souvent à l'échelon mondial. Ainsi, un anticoagulant est fabriqué à partir de saumons

lesquelles un laboratoire n'arrivant pas à honorer ses engagements assume financièrement la charge du surcoût entraîné, ce qui n'est plus le cas dans le cadre d'un contingentement décidé par l'ANSM ? Voilà une première mesure que l'on pourrait prendre ! Une autre question subsiste vise les mesures pour relocaliser en France et en Europe la fabrication des matières premières. Je concède que vous n'êtes certainement pas la seule ministre concernée par ce sujet. À tout le moins, l'ANSM ne pourrait-elle pas imposer aux laboratoires étrangers les normes drastiques qu'elle impose aux laboratoires français ? ministre, la colère monte sur ce sujet et je pense que vous en êtes consciente.

parce qu'ils sont imprononçables pour le néophyte que je suis : « Chaque jour, un nouveau médicament [est] en rupture, c'est la gabegie totale et les labos ne nous informent pas. On se fait engueuler

En 2015, 391 médicaments étaient indisponibles ou en rupture de stock, contre 530 pour l'année 2017. Selon un sondage récent, la moitié des Français a déjà été confrontée à une rupture de stock ou d'approvisionnement en médicament. Dans un cas sur cinq, ces pénuries concernent un vaccin.

Ce problème n'est pas nouveau, mais il a pris une ampleur considérable. Dès 2015, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé alertait sur des orientations dans l'organisation de la production qui pourraient conduire à une explosion du nombre de pénuries. Elle ne s'était pas trompée : les pénuries ont augmenté de 30 % en un an. la Charente-Maritime, environ 4 % des médicaments sont en rupture de stock ou d'approvisionnement. Cette moyenne départementale est quasi équivalente à la moyenne nationale, qui se situe à 5 %. Nous sommes donc bien loin des ruptures anecdotiques occasionnelles du siècle dernier.

ce qui incite certains laboratoires à faire le choix de distribuer leurs médicaments dans des pays étrangers. Pour toutes ces raisons, madame la ministre, je souhaite connaître les actions que le Gouvernement entend mener, afin d'endiguer ces ruptures de stock et ces difficultés d'approvisionnement.

Vous avez raison, le circuit de distribution des médicaments français est régulièrement touché par des dysfonctionnements, qui entraînent de nombreuses ruptures d'approvisionnement en médicaments. En France, le nombre de ruptures et de risques de rupture de médicaments s'est accru de manière significative depuis 2008. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM, indique que les ruptures de stock ont touché près de 530 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur à l'échelon national en 2017, soit une augmentation de plus de 30 % en un an. À titre de comparaison, en 2008, on dénombrait seulement 44 de ces médicaments en situation de rupture, soit plus de dix fois moins.

d'un moment à l'autre conduire à augmenter les besoins en médicaments, si les indications progressent considérablement. En réponse à ces difficultés, la France a mis en oeuvre des mesures de prévention des ruptures. Le mécanisme juridique élaboré, depuis 2016, permet normalement de lutter contre les ruptures d'approvisionnement à l'échelle nationale et de garantir l'accès de tous les patients à leur traitement. Ces dispositions imposent notamment aux titulaires d'autorisation de mise sur le marché et aux exploitants des médicaments d'élaborer et de mettre en oeuvre des plans de gestion des pénuries pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur- je pense notamment aux médicaments anticancéreux - et de les soumettre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. En complément, deux arrêtés des 26 et 27 juillet 2016 ont fixé la liste respectivement des vaccins et des classes thérapeutiques contenant des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur devant faire l'objet de plans de gestion des pénuries.

Au quotidien, chez les répartiteurs comme dans les pharmacies d'officine, nous n'en ressentons pas les effets : nous rencontrons des difficultés pour obtenir des informations de la part des laboratoires, notamment sur les

C'est la conséquence, d'une part, de l'insuffisance des moyens financiers, matériels et en personnel mis à la disposition des EHPAD et, d'autre part, du fait que ces établissements accueillent un nombre croissant de personnes très âgées, souvent grabataires et réclamant de ce fait des soins beaucoup plus importants. Or, si la France est aujourd'hui un pays développé, c'est grâce au travail des générations qui nous ont précédés. À l'époque, on travaillait beaucoup plus que 35 heures par semaine, il n'y avait pas de RTT ni cinq semaines de congés payés. Notre société a de ce fait l'obligation morale de faire tout son possible pour que les personnes âgées auxquelles nous sommes globalement tous redevables soient accueillies et accompagnées dans des conditions matérielles et humaines satisfaisantes. Hélas, ce n'est pas le cas : les gouvernements successifs n'ont pas débloqué les moyens nécessaires. Dans le département de la Moselle,

En effet, à l'époque de la sidérurgie et des houillères, ce département comptait une population jeune, laquelle est aujourd'hui entrée dans le troisième âge. Ayant moins de besoins par le passé, la Moselle avait créé moins de places en EHPAD par rapport au ratio démographique. Le vieillissement accéléré de la population mosellane doit maintenant être pris en compte par un effort de rattrapage. de rattrapage. Madame la ministre, comment envisagez-vous de répondre aux besoins qualitatifs qui existent partout en France et aux besoins quantitatifs propres à certains départements comme la Moselle ?

Ma conviction, depuis maintenant un an, est que notre pays n'a pas encore su trouver un véritable modèle de prise en charge de la perte d'autonomie. L'attente de la société est pourtant légitime. Le vieillissement doit être anticipé et c'est le rôle des pouvoirs publics, au sens large, de préparer l'avenir, d'impulser le changement, de donner un cap. J'ai présenté voilà trois semaines une nouvelle feuille de route et annoncé des moyens supplémentaires. Ainsi, 15 millions d'euros seront alloués en 2018 au financement de plans de prévention en EHPAD. Ces moyens seront portés à 30 millions d'euros à partir de 2019 pour la prévention de perte d'autonomie. 100 millions d'euros seront consacrés à la refonte du mode de financement de l'aide à domicile. Par ailleurs, les EHPAD recevront 360 millions d'euros supplémentaires de 2019 à 2021 pour recruter des personnels soignants. 1 000 places d'hébergement temporaire en EHPAD pour les personnes sortant d'hospitalisation seront financées à hauteur de 15 millions d'euros par l'assurance maladie dès 2019, l'objectif étant de réduire les durées d'hospitalisation et de faciliter le retour à domicile des personnes. Enfin, un effort financier de 40 millions d'euros permettra de généraliser l'accès à la télémédecine en EHPAD. À cela s'ajoute le recrutement d'infirmières de nuit pour couvrir l'ensemble des EHPAD d'ici à 2020. S'agissant plus particulièrement du département de la Moselle, l'agence régionale de santé, conjointement avec le département, a engagé une démarche de rattrapage. Dans le cadre des restructurations hospitalières, un projet médico-social pour la Moselle-Est a été arrêté et a permis de créer 455 places sur les territoires du bassin houiller et de Sarreguemines, dont 163 places en EHPAD et 69 places de services de soins infirmiers à domicile. Dans le secteur de Thionville, le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie 2017-2021 prévoit également la création de 275 places en EHPAD. Je vous confirme donc que la démarche de réajustement en termes d'équipement dans le département de la Moselle se poursuit, tout comme l'évolution et la transformation de l'offre, notamment par le biais des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. La parole

notamment sur une nécessaire adaptation et évolution du tarif des EHPAD, ainsi que sur l'évolution du métier d'aide-soignant et des autres personnels pour adapter ces métiers et les revaloriser. Je souhaite vivement que ces différentes propositions soient prises en compte. La

annuel publié au mois de février dernier, la Cour des comptes rappelle que le coût du déploiement des compteurs Linky est couvert dans « des conditions avantageuses pour Enedis » par les consommateurs, les magistrats relèvent également les insuffisances techniques du compteur. Ils rejoignent en cela les conclusions de l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, laquelle avait déjà alerté sur le fait que les informations auxquelles auront accès les utilisateurs n'étaient ni assez nombreuses ni suffisamment accessibles pour faire du compteur Linky un véritable outil de maîtrise de consommation. En effet, l'affichage déporté, permettant une information en temps réel plus complète et lisible, est limité aux seuls ménages précaires et les portails internet du distributeur et des fournisseurs ne permettent pas une information détaillée et circonstanciée. Comme le mentionnent pourtant les magistrats, « la connaissance par l'usager de sa consommation d'électricité à un [laps] de temps suffisamment court [ ...] constitue un prérequis à la mise en place de toute action de MDE [maîtrise de la consommation d'énergie] à un niveau individuel. Cela étant, dès 2010, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, demandait déjà que le compteur dispose d'un afficheur déporté, solution d'information en temps réel en kilowattheures comme cela a pu se faire ailleurs en Europe, notamment au Royaume-Uni. Le Médiateur national de l'énergie a également plaidé pour la généralisation d'un tel dispositif, réclamé par plus de 150 000 citoyens, qui ont signé une pétition en ce sens. Aussi, madame la secrétaire d'État, je souhaite connaître les dispositions que le Gouvernement compte prendre afin de faciliter réellement l'accès des consommateurs au suivi en temps réel de leur consommation d'énergie et les améliorations qu'il entend apporter au dispositif. La parole

Il permet des opérations à distance, comme la relève des données de consommation. Il permet aussi d'éviter les facturations estimées, qui donnent parfois lieu à des rattrapages importants. Il favorise surtout le développement des énergies renouvelables, l'autoconsommation et améliore la gestion du réseau. En matière de consommation, le compteur Linky peut permettre à chaque consommateur d'avoir une meilleure connaissance de sa consommation électrique, donc de participer à l'objectif de maîtrise de la consommation d'énergie. Ce sont des éléments indispensables pour accélérer la transition énergétique. de participer aux efforts de maîtrise de la demande, chaque consommateur peut accéder à ses historiques de consommation sur le site internet d'Enedis. Il est vrai que des efforts de communication et d'accompagnement additionnels

ce qui est généralement peu lisible pour les consommateurs. Seuls les fournisseurs sont en mesure de faire part de consommations en euros, alors que ces dernières sont plus directement utilisables par le consommateur. Les fournisseurs d'énergie devraient être plus impliqués.

Le gouvernement actuel, comme le précédent, considère qu'il faut favoriser le retour à l'emploi des seniors, ce que doit permettre le plan senior, lancé à l'occasion de la grande conférence sociale de juillet 2014. Or, pour ma part, j'ai reçu de nombreux témoignages de seniors, qui, sortis de l'emploi et malgré une recherche active, ne trouvent pas d'employeurs prêts à les embaucher à un ou deux ans de la retraite. Ils deviennent alors la « cible » de Pôle emploi, qui leur demande de prospecter dans d'autres domaines que celui de leurs compétences, de baisser leurs prétentions salariales, ou encore de suivre des formations pour ne pas être radiés des fichiers. À quelques mois de leur retraite, il n'est ni réaliste ni socialement justifié de leur imposer des actions de recherche active d'emploi ou la participation à une formation inutile et souvent coûteuse. Il conviendrait donc de rétablir la dispense de recherche d'emploi ou, du moins, d'étudier un aménagement de ce dispositif pour les chômeurs seniors proches de la retraite et de permettre, ainsi, à Pôle emploi de concentrer ses forces sur d'autres catégories de demandeurs d'emploi. Par conséquent, je demande au Gouvernement s'il envisage de remettre en place ce dispositif de dispense de recherche d'emploi lors de l'examen du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

C'est pour cela que nous menons une politique volontariste, qui vise à favoriser le développement de l'emploi, notamment l'emploi des seniors, en renforçant les droits des salariés et des demandeurs d'emploi. C'est le sens de la rénovation profonde de notre modèle social que nous avons engagée avec les ordonnances pour le renforcement du dialogue social. La ministre du travail, Muriel Pénicaud, la poursuit à présent avec le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dont le vote en première lecture à l'Assemblée nationale aura lieu cet après-midi. est de créer, pour la première fois, une véritable sécurité professionnelle, universelle, simple et efficace, qui accompagnera chacun tout au long de son parcours professionnel. Dans un monde où 50 % des emplois seront profondément transformés dans les dix années à venir, cela passe par un accès facilité à l'atout majeur du XXI siècle : les compétences. C'est pourquoi, en complément de l'effort sans précédent de 15 le cadre du plan d'investissement dans les compétences, nous transformons le système de la formation professionnelle pour le rendre plus réactif face aux mutations, plus lisible et plus juste. S'agissant spécifiquement de l'assurance chômage, nous expérimenterons un dispositif de « journal de bord Il doit permettre de rendre les démarches de candidatures plus efficaces, de prévenir le découragement et de mieux préparer les entretiens avec les conseillers. C'est par des moyens pragmatiques, qui remettent nos concitoyens au coeur des dispositifs, que nous poursuivrons l'amélioration de l'emploi des seniors, et non par le rétablissement d'une dispense de recherche d'emploi, qui ne ferait qu'accélérer leur retrait du marché du travail. La parole

résultats, je le crains, peu probants. Cela étant, il n'est pas interdit d'espérer, encore moins de réussir

et solidaire. Madame la secrétaire d'État, les conséquences sanitaires de la forte concentration d'industries lourdes dans le golfe de Fos, situé entre le delta du Rhône et l'étang de Berre, doivent retenir toute notre attention. Les élus et les populations concernés entreprennent depuis de nombreuses années d'interpeller l'État à ce sujet. Le bassin industrialo-portuaire de Fos s'étend sur 10 000 hectares et regroupe près de 40 000 salariés au sein de 200 entreprises. On y recense pas moins d'une trentaine de sites classés Seveso. Depuis maintenant quatre décennies, 100 000 habitants sont exposés aux dangers sanitaires qu'une telle activité est susceptible de faire courir. Provence-Alpes-Côte d'Azur, a reconnu que les habitants de Fos-sur-Mer connaissent « un état de santé fragilisé, dans une zone fragilisée par la pollution environnementale Dioxines, benzène, plomb, de récentes études entreprises par le milieu associatif relèvent une surimprégnation des personnes exposées quotidiennement. Élus locaux et parlementaires des Bouches-du-Rhône sont conviés dans une semaine, à Istres, pour la restitution du rapport réalisé par le Conseil général de l'environnement et du développement durable sur la pollution de l'air dans ce secteur. Madame la secrétaire d'État, le Gouvernement peut-il s'engager à poursuivre ce travail d'évaluation, en liaison étroite avec la population, afin de faire valoir

Comme vous le mentionnez à juste titre, la zone de Fos-étang de Berre est l'une des plus importantes concentrations industrielles en France et les pollutions d'origine industrielle, résidentielle ou liées aux transports s'y cumulent. Je tiens à vous

de l'été. Malgré la réduction des émissions industrielles ces dix dernières années, les efforts doivent absolument être poursuivis. C'est pourquoi nous avons demandé au préfet d'établir, en liaison avec les industriels concernés, un plan de réduction des émissions industrielles. Par ailleurs, comme vous le savez, l'Association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos a réalisé une étude sur les produits AOC du département, à partir de prélèvements effectués entre 2009 et 2015. Elle conclut dans son rapport que des polluants sont détectés dans les denrées alimentaires d'origine animale animale produites à proximité de la zone industrielle du golfe de Fos et que les résultats obtenus sont imputables à l'activité industrielle présente. Il y a donc un lien avéré. Mais sur l'ensemble des échantillons prélevés et analysés, seuls deux résultats dépassent les teneurs maximales réglementaires. Par ailleurs, les services du ministère de l'agriculture ont réalisé en 2017, dans le cadre des plans de surveillance et des plans de contrôle, quarante prélèvements de recherche dans des denrées alimentaires. Tous les résultats obtenus se sont révélés conformes aux teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires. Néanmoins, aucun risque à l'égard de ces populations ne doit être négligé, nous en sommes bien conscients, madame la sénatrice. Une nouvelle campagne de prélèvements et d'analyses sera donc réalisée à proximité des installations industrielles du golfe de Fos. À cet effet, nous avons saisi l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement

ce qui se traduirait à l'échelle de la France par 500 postes supprimés et une baisse de 2 % du budget. Cela ne sera pas sans effet sur les centres ouverts restants, comme celui de Lyon-Bron, qui devra non seulement endosser les missions et l'activité des établissements fermés, mais aussi le faire avec un budget et des effectifs en baisse. Les personnels du centre de Lyon-Bron sont inquiets de devoir, à l'avenir, concentrer toute l'activité météorologique régionale. Seront-ils en capacité de remplir leur mission ?

Il faut rappeler que les analyses produites par Météo-France sont des données très utilisées par les différents acteurs locaux : agriculteurs, entreprises, collectivités. Madame la secrétaire d'État, à la lumière de l'exemple lyonnais, pouvez-vous nous préciser les intentions du Gouvernement concernant le devenir de Météo-France et, plus généralement, les orientations qu'il souhaite donner au plan Action publique 2022 ?

maîtriser les dépenses publiques, en optimisant les moyens des administrations et des opérateurs de l'État. C'est tout l'objet du programme Action publique 2022, que vous avez mentionné. C'est pourquoi le Gouvernement a demandé au président-directeur général de Météo-France d'élaborer un projet global concernant l'établissement. Par ailleurs, les progrès en matière de modélisation numérique du temps doivent permettre de consolider la finesse des prévisions météorologiques et climatiques, notamment pour ce qui concerne les zones de relief. Pour permettre leur intégration dans la prévision opérationnelle, il est donc prévu de conforter les moyens de calcul de haute performance de l'établissement, qui s'est également traduit budgétairement. Cela permettra notamment une meilleure anticipation des risques sur les territoires de montagne. Le contrat d'objectifs et de performance 2017-2021 de l'établissement confirme d'ailleurs cette orientation. Il propose, pour les activités de sécurité des personnes et des biens et de prévision généraliste, une structuration du réseau territorial de Météo-France en métropole autour de sept centres météorologiques interrégionaux. Ainsi, les activités de climatologie et de prévision sur le Cantal, la Drôme et le Puy-de-Dôme seront progressivement reprises à l'échelle interdépartementale, et les ressources de Météo-France à terme concentrées au sein du centre interrégional de Lyon-Bron. Nous veillerons à la poursuite, par Météo-France, de la conduite des évolutions du réseau territorial lui permettant de remplir ses missions en conservant une qualité de service optimale, tout en tenant compte de l'évolution de ses effectifs, de ses besoins et des moyens technologiques. Telle est l'équation que nous voulons résoudre.

je veux vous rappeler que le Sénat n'a eu de cesse d'appeler l'attention du Gouvernement sur la dégradation de la cohésion des territoires. J'espère que ce dernier saura s'en souvenir lorsqu'il mettra en place le plan Action

au travail Bourgogne-Franche-Comté impose aux maîtres d'ouvrage de bâtiments et à leur maître d'oeuvre l'installation de garde-corps permanents et non rabattables au niveau des accès et périphéries de la totalité des toitures planes. Or le code du travail prévoit que la prévention des chutes de hauteur est assurée soit « par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée », soit « par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente. Il n'existe donc aucune obligation légale d'installer des garde-corps permanents et non rabattables, comme l'exige la caisse régionale. La Cour de cassation l'a d'ailleurs rappelé récemment dans une jurisprudence claire. Pourtant, les acteurs du bâtiment qui utilisent des garde-corps rabattables se voient opposer un refus catégorique et systématique de la part de la CARSAT ou, plus précisément, de l'un de ses agents, sans doute trop zélé. Ils sont alors soumis à une procédure de majoration de leur taux de cotisation, qui peut s'élever jusqu'à 200 %, et à d'autres sanctions financières insupportables, notamment pour les collectivités. vous comprendrez donc tout l'enjeu de ma question. Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer précisément si le recours à des garde-corps rabattables, ou à tout autre dispositif de sécurité équivalent, est conforme ou non à la réglementation relative au travail en hauteur. Si le Gouvernement l'estime ainsi, comme l'a jugé la Cour de cassation,

matin. Je vous remercie de cette question, qui touche à un sujet important pour la santé et la sécurité au travail, celui de la prévention des risques liés au travail en hauteur. est la troisième cause d'accidents du travail mortels, responsable de 13 % des décès sur les 514 accidents du travail mortels recensés en 2016. Comme vous le savez, les risques de chutes de hauteur font l'objet d'une attention toute particulière, parce qu'ils font partie des risques prioritaires dans le cadre du troisième plan santé au travail. L'objectif est clairement de faire progresser la prévention des chutes, en faisant évoluer les pratiques des acteurs de l'entreprise et de la construction, pour réduire le nombre et la part des accidents du travail dus aux chutes. Concernant les moyens d'intervention des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, le code de la sécurité sociale prévoit qu'elles peuvent « inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention ». ces dispositions, le réseau des CARSAT se voit conférer un large pouvoir de recommandation et d'injonction, sans le support d'aucune prescription réglementaire puisqu'il peut donc prescrire des mesures ne figurant pas expressément dans le code du travail à partir du moment où elles contribuent à la prévention, comme l'a précisé le Conseil d'État voilà plus de vingt ans. En l'espèce, la CARSAT régionale est fondée à imposer aux acteurs de la construction les mesures de prévention qu'elle a jugées appropriées. Car les dispositions du code du travail relatives à la prévention des chutes de hauteur donnent justement une marge d'appréciation aux employeurs et préventeurs,

Je pense également au ferroutage et vous interroge sur les suites et le calendrier de l'appel à manifestation d'intérêt public, lancé en avril 2018. Je pense enfin à la réouverture de la ligne ferroviaire Pau-Canfranc-Saragosse, cheval de bataille du président Alain Rousset. ces solutions, si pertinentes soient-elles, ne dévieront qu'une part réduite du trafic de l'A63. C'est pourquoi je souhaite insister de nouveau sur la nécessité de solutions alternatives routières transpyrénéennes. Un axe potentiel existe à l'est du département des Pyrénées-Atlantiques. En effet, le pôle Pau-Oloron-Sainte-Marie, alors qu'il fait preuve d'un dynamisme économique avéré, est isolé, car sans raccordement digne de ce nom à l'Espagne, notamment à la région de Saragosse. Au contraire, l'Espagne a construit un réseau routier : il relie Saragosse au Somport, mais débouche malheureusement, côté français, sur la route nationale 134, qui n'est pas à la hauteur des trafics actuels et encore moins de Il y a donc urgence à moderniser la route nationale 134, à réaliser l'évitement des bourgs et l'élargissement de certains tronçons. Cela permettrait d'ouvrir un itinéraire vers le centre de la France, en direction de Limoges, délestant à terme le trafic supporté sur l'axe Hendaye-Bordeaux. Cette sécurisation de la route nationale 134, en particulier les déviations de villages, doit être envisagée à un horizon raisonnable. Cela n'exclut pas la réalisation, à plus long terme, d'une voie rapide entre

Élisabeth Borne ne pouvant être présente ce matin, elle m'a chargée de vous répondre. L'État est conscient des enjeux de sécurité et d'environnement liés au trafic routier. C'est pour cela qu'il s'efforce d'adapter et de moderniser le réseau au sud de Bordeaux. La section centrale de l'A63 et la section entre Ondres et Biarritz ont notamment été aménagées, mises à deux fois trois voies et aux normes autoroutières. De plus, la section entre Biarritz et Biriatou est actuellement en travaux, pour une mise en service effective prévue au cours du second semestre de Par ailleurs, la modulation des tarifs de péage autoroutiers, en fonction de la norme euro des véhicules, appliquée sur la section centrale de l'A63 constitue une incitation supplémentaire à la modernisation des flottes de poids lourds. Au-delà, vous savez que la France est engagée, aux côtés de l'Espagne, pour limiter les trafics de poids lourds sur les axes routiers pyrénéens. Un accord a d'ailleurs été conclu en 2009 pour développer deux services d'autoroute de la mer sur la façade atlantique. La France et l'Espagne collaborent aussi depuis 2015 en vue d'instaurer des services d'autoroute ferroviaire sur les versants atlantique et méditerranéen des Pyrénées. Pour finir, monsieur le sénateur, je rappelle qu'un appel à manifestation d'intérêt auprès des constructeurs de matériel roulant a eu lieu en 2017. pour optimiser les conditions de développement de nouveaux services de ce type, un appel à manifestation d'intérêt commun avec l'Espagne, notamment sur l'axe atlantique, est en cours. Les réponses sont attendues pour la fin du mois de juillet, donc très prochainement. La parole

que la course ne soit perdue d'avance, car la mise à deux fois trois voies ne répond pas finalement, à terme, à l'augmentation très forte du trafic, essentiellement routier. Dans vos propos, je reconnais la volonté du Gouvernement de développer le ferroutage. J'avais moi-même mentionné cet appel à manifestation d'intérêt et les autoroutes de la mer, même si je pense que peut être développée davantage encore cette branche de l'alternative au transport routier. J'ai en revanche des réticences par rapport à ce que vous avez dit sur la volonté de ne pas développer d'autres axes routiers transpyrénéens. Il y a un axe qui peut se dessiner

et du ferroutage, la nécessité de sécuriser la route nationale 134 et de penser vraiment à une liaison entre Pau, Oloron et Le Somport, susceptible de préfigurer une prolongation vers le centre de la France et Limoges.

Alors qu'un certain nombre de projets sont reportés, le COI confirme dans son rapport l'utilité et la nécessité des infrastructures structurantes que sont les LGV Bordeaux-Toulouse et Montpellier-Béziers-Perpignan. À présent, l'enjeu est leur réalisation dans des délais qui répondent aux besoins et à l'attente de nos concitoyens. Les pistes de financements nouveaux, portées par les collectivités concernées auprès du Gouvernement, sont en grande partie reprises dans les préconisations du COI. L'équation est maintenant non plus technique ou financière, mais bien politique, ce qui renvoie aux choix que devront faire dans les prochaines semaines le Gouvernement et les parlementaires dans le cadre du futur projet de loi d'orientation sur les mobilités. La LGV Bordeaux-Toulouse comme la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan doivent s'inscrire dans le scénario 3, le plus volontariste, figurant dans le rapport. Alors que le COI appelle à un aménagement du territoire équilibré et à une plus grande équité, je souhaite que ces choix politiques prennent en compte les grandes difficultés de déplacement des 6 millions d'habitants de l'Occitanie, région la plus dynamique de France en termes d'emplois et d'habitants. Je souhaite également connaître les intentions du Gouvernement pour mettre fin à cette situation vieille de vingt-cinq ans. La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.

Je ne peux que me ranger à votre avis. La ligne Bordeaux-Toulouse est un projet essentiel pour répondre durablement aux besoins de mobilité des Français. Priorité doit être donnée aux aménagements des noeuds ferroviaires de Bordeaux et de Toulouse, qui constituent un préalable indispensable à la réalisation de la ligne nouvelle. Cela permettra aussi de redonner de la régularité au transport du quotidien, qui est, vous le savez, une priorité de ce gouvernement. Le projet de ligne nouvelle Montpellier-Perpignan doit, quant à lui, répondre à la demande croissante de mobilité et aux problèmes de congestion qui en découlent sur l'axe ferroviaire du Languedoc-Roussillon. Il permettra aussi de créer un service à haute fréquence et d'assurer, à terme, la continuité de la grande vitesse ferroviaire entre la France et l'Espagne. Comme vous le savez, madame la sénatrice, le principe d'une réalisation phasée de la ligne nouvelle a été La première étape sera la liaison mixte, fret et voyageurs, entre Montpellier et Béziers. Ces lignes nouvelles, Bordeaux-Toulouse et Montpellier-Béziers, représentent un investissement total de près de 8 milliards d'euros. son rapport, le COI préconise d'engager ces opérations dans la période 2018-2022 et la première phase Toulouse-Agen dans la période 2028-2032. Ce calendrier devrait être mis en regard avec des ressources qui pourraient être mobilisées en tenant compte des besoins de remise à niveau des réseaux existants.

Madame la secrétaire d'État, l'enjeu principal pour développer un territoire et attirer de la main-d'oeuvre, c'est la mobilité grâce au développement des axes de transport. C'est particulièrement vrai dans les territoires ruraux. Dans les Pays de la Loire, plusieurs projets structurants ont été mis soit au tapis, soit à l'arrêt. L'abandon par l'État de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a été une douche froide. L'attractivité du Grand Ouest reposait entre autres sur ce grand projet d'aéroport.

lancé en 2006 par Laval agglomération et par le département de la Mayenne, afin de renforcer la compétitivité et l'attractivité du territoire, notamment dans le secteur de la logistique. Situé sur les communes d'Argentré et de Bonchamps-lès-Laval, ce parc comporte trois axes majeurs : la création d'une zone d'activités, un accès direct à l'autoroute A81 et un embranchement ferré. Il s'agit d'un projet d'envergure industrielle et d'aménagement du territoire. Il prévoit en effet une desserte assurée par un nouveau point d'échange sur l'autoroute A81. La création de cette nouvelle infrastructure est primordiale pour la réussite du parc. L'échangeur a été retenu dans le plan d'investissement autoroutier décidé en 2016 par le Président de la République. Cette inscription prenait acte d'une participation financière de l'État à hauteur de 1,4 million d'euros, sur un total de 9,6 millions

S'engager avec fermeté et responsabilité sur des projets locaux comme celui-ci permet de désenclaver les territoires ruraux comme le mien. Ma question est la suivante : l'État soutient-il le projet de parc de développement mayennais, avec sa connexion directe au réseau autoroutier ?

Monsieur le sénateur, je le répète, Élisabeth Borne ne pouvant être présente ce matin, elle m'a chargée de vous répondre. Dans le cadre du projet de loi d'orientation sur les mobilités qu'Élisabeth Borne présentera ici cet été, soyez assuré que le Gouvernement veillera à proposer des solutions de mobilité adaptées adaptées à tous les territoires, en particulier à ceux qui ont besoin d'être désenclavés et d'être reliés au réseau principal. S'agissant du réseau routier national non concédé desservant les territoires ruraux, les moyens consacrés dans l'actuel contrat de plan État-région aux axes desservant les villes moyennes et les territoires ruraux

ont mis en évidence la nécessité de faire porter en priorité les efforts sur la remise à niveau du réseau et sur la désaturation des noeuds ferroviaires. Par ailleurs, le Gouvernement s'est engagé à ne pas suivre les recommandations du rapport Spinetta sur le sujet dit des « petites lignes ». L'État demeurera aux côtés des collectivités pour maintenir ce réseau. Quant aux engagements qu'il a pris au titre des contrats de plan État-région, ils seront tenus. Concernant les projets du Grand Ouest, à la suite de la décision prise par le Premier ministre sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le Gouvernement a lancé une concertation avec les élus des territoires Une mission est actuellement conduite par M. Francis Rol-Tanguy, visant à faire émerger un pacte d'accessibilité pour la Bretagne et un contrat d'avenir pour les Pays de la Loire. M. Rol-Tanguy remettra son rapport dans les prochains jours et, sur cette base, Élisabeth Borne formulera des propositions pour la programmation des grandes infrastructures de transport du Grand Ouest. Vous voyez que nous sommes actifs sur cette question et que de nombreuses décisions seront prises prochainement. D'autres seront débattues ici. La parole

madame la secrétaire d'État, d'y répondre. Alors que les troupeaux rejoignent les alpages, notamment dans les Alpes du Sud, je souhaite avoir des précisions sur le plan national d'actions 2018-2023 sur le loup et les activités d'élevage qui prévoit la mise en place d'une série de mesures visant à contenir la population lupine dans le but de préserver l'activité d'élevage et le pastoralisme. C'est la raison pour laquelle, dans les départements concernés par les dommages causés par le loup, comme dans celui des Hautes-Alpes, une équipe de louvetiers est requise. Ces lieutenants de louveterie, nommés par le préfet, sont placés sous son autorité pour réaliser des missions d'ordre public

avec du matériel adapté, par exemple des caméras thermiques. Aussi, afin de soutenir l'action des louvetiers, je vous serais reconnaissante de bien vouloir m'indiquer si des crédits seront mis à disposition des préfets. Dans l'affirmative, je vous remercie également de bien vouloir me préciser sur quelle enveloppe ils seront mobilisés. La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire. Madame la sénatrice Patricia Morhet-Richaud, je vous réponds à la place du ministre de l'agriculture et de l'alimentation et du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, aucun d'entre eux n'ayant pu être présent aujourd'hui, ce qu'ils regrettent.

Son objectif fondamental est de concilier préservation de l'espèce et maintien du pastoralisme. C'est un équilibre difficile. Un programme de soutien du pastoralisme vise donc à améliorer la protection des troupeaux et à faciliter leur défense en cas d'attaques. Les mesures de protection seront financées à 80 % et un observatoire pour le suivi de leur mise en oeuvre sera créé. Des expérimentations seront mises en place dans les territoires volontaires et un réseau technique « chiens de protection » sera développé. Le Gouvernement vient d'ouvrir les crédits nécessaires aux premières expérimentations de bergers mobiles dans des parcs nationaux. Face à la persistance de la prédation dans certaines zones, malgré le déploiement des mesures de protection, la politique d'intervention sur les loups a été modifiée pour faciliter la défense des troupeaux. Les tirs de défense réalisés à proximité des troupeaux peuvent être effectués toute l'année, par la brigade nationale « loup

Le plan prévoit par ailleurs une action spécifique pour accompagner les actions des louvetiers auprès des éleveurs, tant pour les tirs de défense que pour les tirs de prélèvement. Les louvetiers sont amenés à effectuer de nombreux déplacements pour soutenir des bergers et des éleveurs confrontés à des attaques. Ils sont tous bénévoles et travaillent donc sans percevoir de rémunération. Cependant, je vous confirme qu'un budget de 142 000 euros vient d'être mis à disposition afin de leur verser des indemnités kilométriques et de leur fournir un matériel adapté, tel que des caméras thermiques, pour remplir leur mission, notamment la nuit. Le Gouvernement a ainsi mis en place une dynamique qui permettra de soutenir les éleveurs confrontés à la prédation et d'optimiser l'action des différents acteurs présents sur le terrain, qu'il s'agisse des bergers ou des lieutenants de louveterie.